Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la mission « Économie » porte un ensemble de dispositifs en faveur des entreprises, et notamment des PME dans les secteurs de l'artisanat, du commerce et de l'industrie. La mission porte aussi sur les crédits des administrations, autorités administratives indépendantes et opérateurs chargés de la mise en oeuvre de ces politiques, ainsi que ceux de l'Insee et des services économiques du Trésor à l'étranger.

cette augmentation résulte principalement de la très nette croissance des crédits consacrés au dispositif de compensation carbone des sites électro-intensifs, à savoir 173 millions d'euros, soit une hausse de 160 %. En dehors de cette mesure, les moyens des trois programmes « permanents » de la mission sont globalement en baisse. La plus grande partie de l'effort de baisse repose sur les différents dispositifs de soutien à l'activité des entreprises. Entre 2014 et 2020, le montant total de ces dispositifs a été considérablement considérablement réduit, passant de 234 millions d'euros en 2014 à 68 millions d'euros en 2020, soit une baisse de 71 %. La « rationalisation » des dispositifs de soutien se résume trop souvent une logique de « rabot », année après année. Or cette érosion ne fait pas une politique. En fin de compte, les réductions proposées ne donnent pas vraiment de sens à la politique et aux choix qui sont faits. La dernière victime de cette politique de rabot a été le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (Fisac), placé en « gestion extinctive » depuis le 1 janvier dernier. Après avoir vu sa dotation passer de 78 millions d'euros en 2010 à seulement 16 millions d'euros en 2018, le Fisac a été placé en gestion extinctive à partir de cette année. En clair, il a été supprimé, avec seulement 2,8 millions d'euros de crédits de paiement pour 2020 destinés à couvrir les opérations décidées avant 2019. Je présenterai tout à l'heure un amendement visant à réabonder le fonds en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, afin de permettre de mobiliser de nouveau cet outil en direction des territoires les plus fragiles. d'exonération des commerces en fiscalité locale offerte aux collectivités ne suffira pas, à elle seule, à pallier la disparition de cet effet de levier indispensable pour les territoires. Plus globalement, la logique sous-jacente à l'évolution de la mission « Économie » est celle d'un désengagement progressif de l'État en matière de soutien aux petites entreprises, aux commerçants, aux artisans. Le message est le suivant : c'est le rôle des collectivités locales, et surtout celui des régions depuis la loi NOTRe de 2015. Je voudrais néanmoins, madame la secrétaire qu'à titre exceptionnel vous avez su être présente, notamment à l'occasion du G7, pour accompagner les commerçants qui se sont vu indemniser. Je dois souligner la réactivité et l'efficacité qui a été la vôtre sur ce dossier. J'en viens maintenant aux administrations de la mission. Là aussi, l'effort est important, puisque 267 postes seront supprimés en 2020 sur le périmètre de la mission, dans le cadre d'un « recentrage » sur certaines actions prioritaires.

poursuivra quant à elle la rationalisation de son réseau à l'étranger, avec la suppression de 40 ETP en 2020. Entre 2009 et 2018, l'effectif des services à l'étranger est ainsi passé de 1 339 à 622 agents, soit une baisse de 54 %. Je terminerai par quelques mots sur le plan France Très haut débit. Le programme 343, qui lui est consacré, porte la participation de l'État, soit au total 3,3 milliards d'euros, afin d'assurer la couverture de 100 % du territoire d'ici à 2022. Sur le plan budgétaire, les crédits annoncés sont là, l'échéancier suit son cours et 440 millions d'euros de crédits de paiement sont prévus pour 2020. Sur le terrain, en revanche les choses sont plus complexes. Seuls 36 % des locaux situés dans les zones les moins denses sont à ce jour éligibles à la fibre optique, contre 85 des locaux dans les zones très denses, donc plus rentables. Les causes de ces retards ne sont pas nouvelles et peuvent se trouver à toutes les phases des projets. À mon sens, la priorité doit être accordée à la couverture d'un maximum de locaux, plutôt qu'au déploiement de la technologie la plus performante. Pour cette raison, je tiens à saluer comme une avancée la création, en 2019, d'un « guichet cohésion numérique » doté de 150 millions d'euros pour financer des technologies alternatives- 4G fixe, satellite -dans les zones où la fibre optique ne peut être déployée. L'annonce de la réouverture du guichet d'initiative publique, à hauteur de 140 millions d'euros en autorisations d'engagement, va également dans le bon sens en permettant aux collectivités de cofinancer de nouveaux projets de raccordement au réseau. Il conviendra toutefois d'être très vigilant : cette solution transitoire est louable dans l'immédiat, mais ne doit pas non plus compromettre l'objectif de raccordement à la fibre optique de l'ensemble du territoire au-delà de 2022.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, il est bien plus facile d'être procureur qu'avocat de la défense quand on s'exprime Cela fait maintenant cinq ans que je rapporte ce budget et je dois constater que la politique des gouvernements successifs pour maintenir l'activité des PME et des TPE sur les territoires mérite quand même de ne pas être soulignée. Je vous invite à garder à l'esprit que, lorsqu'il disparaît 30 emplois dans une commune de 3 000 habitants, l'impact est bien plus important que lorsqu'il disparaît 300 emplois dans une ville de 30 000 habitants. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de régénérescence possible. La disparition d'une TPE ou d'une petite PME dans un territoire déjà désertifié va entraîner une amplification de cette désertification.

S'agissant du compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », le Gouvernement a présenté un amendement à l'Assemblée nationale créant un nouveau programme destiné aux prêts octroyés dans le cadre du programme d'investissements d'avenir doté de 200 millions d'euros en autorisations d'engagement et de 100 millions d'euros en crédits de paiement. En 2020, cette opération permettra d'octroyer un prêt de 200 millions d'euros à la société Soitec, dont 100 millions d'euros seront débloqués dès 2020. Ce prêt permettra à l'entreprise de maintenir en France son activité de production de semi-conducteurs. L'intervention de l'État était nécessaire, car il s'agit d'une question de souveraineté. De plus, la création d'un programme au sein de ce compte de concours financiers est neutre d'un point de vue budgétaire. Si le Gouvernement

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, mon propos sera essentiellement centré sur les dispositions de ce budget qui concernent le volet commerce et artisanat. Les crédits consacrés à ces secteurs sont malheureusement de moins en moins importants et de plus en plus dispersés. La politique menée par le Gouvernement en faveur de ces secteurs perd en lisibilité. Alors qu'il existait jusqu'en 2018, au sein du programme 134, « Développement des entreprises et régulation », une action spécifique « commerce, artisanat et services », celle-ci a été rassemblée dans l'action n° 23, Industrie et services, ce qui complique le suivi de cette politique publique. En outre, deux changements sont intervenus au détriment du commerce et de l'artisanat entre 2019 et 2020. Le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce, qui est en gestion extinctive depuis 2019, devrait disparaître définitivement à partir de 2020. Alors qu'il intervenait à hauteur de 70 millions d'euros il y a dix ans, seuls 2,8 millions d'euros de crédits de paiement sont demandés au titre de 2020. Nos territoires vont donc se voir amputer d'un dispositif très utile, qui a fait ses preuves, et qui a longtemps financé jusqu'à mille projets par an de soutien et de revitalisation du commerce et de l'artisanat. Le Gouvernement soutient que le programme Action coeur de ville et les régions prendront désormais le relais du Fisac. Or « Action coeur de ville » ne concernera que 222 villes, essentiellement des villes moyennes et non pas des bourgs en zone rurale. Si les régions bénéficient certes de la compétence économique, elles disposent de moyens limités pour cela. L'abandon sans concertation d'un outil qui a fait ses preuves et dont le Sénat avait souhaité, en outre, faire l'un des éléments de la reconquête commerciale des centres-villes, dans le cadre du pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, ne peut recevoir notre assentiment. Je vous proposerai donc un amendement afin d'ouvrir des crédits pour 2020 dotant le Fisac de 30 millions d'euros. Par ailleurs, le Gouvernement a décidé de revoir les modalités de son soutien en faveur des métiers d'art et du patrimoine vivant et de l'artisanat. Il est ainsi prévu que l'Institut national des métiers d'art (INMA) reprenne certaines des missions de l'Institut supérieur des métiers (ISM). La direction générale des entreprises nous indique viser un autofinancement total de la structure d'ici à 2022. 2022. Dans ce cas, pourquoi tarir ce financement dès 2020 ? Ces métiers contribuent pourtant au maintien et au rayonnement d'un savoir-faire rare, ainsi qu'à la promotion de l'excellence française. Je vous proposerai donc d'ouvrir des crédits afin de pérenniser en 2020 l'action de l'Institut national des métiers d'art en le dotant, comme l'an dernier, de 2,25 millions d'euros. La commission des affaires économiques émet un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission, sous réserve du vote des amendements qui vont vous être proposés. La parole

avis. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, peu de changements s'agissant du volet numérique et postes de la mission « Économie », sur laquelle la commission a émis un avis favorable, mais un acte majeur : la réouverture du guichet France Très haut débit, pour lequel notre commission propose un ajustement. quelques mots rapides sur les avancées en matière d'infrastructures numériques. L'objectif du « bon haut débit » pour tous, soit 8 mégabits par seconde, promis par le Président pour 2020, se met seulement en marche. Ce guichet « cohésion numérique », permettant de recourir aux technologies dites « alternatives », devrait verser en effet les premières aides en cette fin d'année, soit deux ans après son annonce. Aucun suivi n'est précisé quant au déploiement de ces solutions alternatives. Ce qui pose question sur l'opérationnalité ! Concernant le très haut débit pour tous en 2022, soit 30 mégabits par seconde, de gros efforts sont fournis par les opérateurs. Ainsi, de bonne dernière de l'Union européenne en 2018, la France devrait regagner des places avec un déploiement, en fibre, qui dépasse les quatre millions de prises en 2019, contre moins de trois en 2017. Les industriels sont donc au rendez-vous, et il convient de saluer leurs efforts. Mais le plus dur reste à faire : si les grandes villes sont couvertes à 85 % et les villes moyennes à 53 %, les zones rurales, les plus difficiles à couvrir en raison de la dispersion de l'habitat, le sont seulement à 15 %. Il y a donc de quoi s'interroger sur l'après-2022 : comment seront couverts ces territoires ruraux ? Par quelle technologie ? Certaines collectivités ont d'ores et déjà choisi l'option des procédures Amel, en quelque sorte du partenariat public-privé. D'autres privilégient les réseaux d'initiative publique (RIP), mais elles ont besoin de visibilité pour répondre à l'attente des populations et des entreprises. le Gouvernement nous propose de rouvrir ce guichet pour financer de nouveaux RIP. Nous nous en félicitons, mais il le fait au compte-gouttes en recyclant d'anciennes autorisations d'engagement et sans crédits nouveaux, de sorte que le compte n'y est pas. C'est pourquoi, madame la secrétaire d'État, nous vous suggérons d'adresser un message clair aux Français et aux entreprises qui ne sont pas encore couverts par la fibre en abondant les crédits inscrits sur cette ligne à la hauteur des besoins réels. Je reviendrai sur cet amendement lors de son examen. Pour conclure, je poserai deux questions rapides. rapides. En matière de déploiement de la 5G, il est crucial que la France ne prenne pas de retard. Les opérateurs ont besoin de la publication des textes d'application d'août dernier. Où en êtes-vous, madame la secrétaire d'État ? Lors des débats parlementaires, vous nous affirmiez que le processus devrait être rapide. être rapide. Concernant l'avenir de l'internet des entreprises, après les premiers pas prometteurs de l'entreprise Kosc Telecom, ouvrant le marché à la concurrence, voilà que cette dernière risque de mettre la clé sous la porte faute, semble-t-il, de respect des engagements de ces fournisseurs, également concurrents. Sa reprise semble poser également problème. Ne craignez-vous pas, madame la secrétaire d'État, que cette dispersion ne mette à mal l'écosystème dynamique et surtout particulièrement souple et adaptable qui s'était mis en place ces derniers mois à la grande satisfaction de l'ensemble des PME ? La parole est à M.

Parmi ses quatre programmes, une seule action concerne désormais l'industrie. Certes, celle-ci est principalement consacrée à la compensation carbone des électro-intensifs, absolument nécessaire à la sauvegarde de leur existence et de leur compétitivité, face à la multiplication par quatre du prix du carbone en cinq ans. La sanctuarisation des crédits de la compensation carbone fonde l'avis favorable de notre commission. Je m'inquiète, néanmoins, de la tendance globale à la réduction des crédits de la mission « Économie ». Hors compensation carbone, le budget dédié à l'industrie baisse cette 5 %. D'abord, la fuite des crédits se poursuit, avec leur transfert vers les PIA ou vers le fonds pour l'innovation et l'industrie (FII), pour l'instant fantôme. La vigilance du Parlement est requise : d'année en année, la lisibilité de la politique industrielle se réduit, rendant notre contrôle très très difficile. Des lignes budgétaires sont de nouveau supprimées cette année. En particulier, pour le deuxième budget consécutif, le Gouvernement veut éteindre le financement par dotation des activités de garantie bancaire de Bpifrance. Pourtant, celles-ci sont orientées à 90 % vers des TPE françaises dont l'accès au crédit reste limité. Plus de 60 000 entreprises en bénéficient chaque année. le Gouvernement admet lui-même dans les documents budgétaires que les crédits consacrés spécifiquement aux PME industrielles sont de 0 million d'euros pour 2020 La commission des affaires économiques souhaite redonner de l'ambition à la politique industrielle. D'une part, nous proposons de restaurer les crédits dédiés à Bpifrance, dans son rôle d'accompagnement du tissu des entreprises, soumis aux aléas de la conjoncture économique. Nous avons, d'autre part, souhaité, en seconde partie du projet de loi de finances, mieux accompagner la transition environnementale et écologique de notre industrie. C'est un « mur d'investissement » qu'il faut mettre en place pour « verdir » notre outil productif. Les dirigeants de PME sont souvent bien seuls. Le Gouvernement doit aussi développer une véritable vision prospective et stratégique, afin d'accompagner l'évolution des filières, notamment celle du plastique ou du diesel, face à des défis sans précédent. Je voudrais enfin dire un mot du débat qui s'annonce autour de la fiscalité de production. Alors que le Gouvernement prépare pour 2020 un « pacte productif », le taux de taxation de l'industrie française est sept fois supérieur à celui de

que la réforme des impôts de production pèse sur les ressources des collectivités locales, déjà très sollicitées par la suppression de la taxe d'habitation. Il nous faut des garanties fermes en ce sens et une compensation à l'euro près sera le préalable à tout débat serein. Le mieux, c'est que nous ayons des ressources dynamiques, et en aucun cas

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la commission des lois a examiné les crédits du programme 134, « Développement des entreprises et régulations », au titre de ses compétences en matière de droit commercial et de droit de la consommation. Ce projet de budget témoigne de la volonté du Gouvernement de recentrer l'action de l'État en matière de développement économique sur un nombre restreint de priorités, au prix d'un désengagement de certains secteurs de l'économie et de l'assèchement de plusieurs dispositifs de soutien aux entreprises. les moyens dévolus par l'État à ses missions régaliennes de régulation concurrentielle des marchés et de protection des consommateurs sont à peu près consolidés. La commission des lois a été sensible au fait que le souci de maîtriser la dépense publique se traduise au sein de ce programme par une politique de rabot, mais par des choix et des efforts de réorganisation : une fois n'est pas coutume, madame la secrétaire d'État, et c'est tant mieux. Il est heureux que l'État accepte enfin de tirer les conséquences des lois de décentralisation et de supprimer des doublons coûteux pour les finances publiques. Encore faut-il que les autres acteurs publics chargés du développement économique aient les moyens de prendre le relais de l'action de l'État. Ce n'est malheureusement pas le cas. Les chambres de commerce et d'industrie subissent une nouvelle baisse sévère de leurs recettes fiscales. Concernant les régions, les 128 millions d'euros supplémentaires qu'elles tireront du dynamisme de la TVA ne suffiront pas à couvrir l'ensemble des charges nouvelles qui leur sont transférées. La commission des lois craint en particulier que l'extinction progressive du Fisac n'ait des conséquences très préjudiciables pour l'artisanat et le petit commerce, sans que les régions puissent intégralement compenser le retrait de l'État. C'est pourquoi elle a déposé, comme les commissions des finances et des affaires économiques, un amendement tendant à rehausser à 30 millions d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement destinés au Fisac. Dans le domaine de la régulation concurrentielle des marchés et de la protection des consommateurs, la commission des lois reste préoccupée par la diminution du volume des contrôles diligentés par les administrations compétentes

Enfin, la commission a dressé un bilan d'étape de la mise en oeuvre du nouveau régime d'installation des professions réglementées du droit, issu de la loi du 6 août 2015. que l'Autorité de la concurrence s'était fondée sur une méthodologie rigoureuse pour proposer une cartographie des zones d'installation. Toutefois, il apparaît à la commission, d'une part, que le risque d'une dépréciation excessive de la valeur patrimoniale des offices existants n'a pas été entièrement écarté à moyen et long terme, d'autre part, que la procédure de nomination dans les nouveaux offices reste beaucoup trop lourde. L'Autorité de la concurrence a formulé de nombreuses propositions de simplification qui n'ont pas encore été prises en compte intégralement. Certaines d'entre elles nécessiteront d'ailleurs l'intervention du législateur. Il faudra rouvrir ce dossier., au vu de ces observations, la commission des lois a donné un avis favorable à l'adoption des crédits de ce programme, sous réserve de l'adoption de son amendement n° II-515. Mes chers Mes chers collègues, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque unité de discussion comprend le temps de l'intervention générale et celui de l'explication de vote. Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de dix minutes pour intervenir. Dans la suite de la discussion, la parole est à M. Xavier Iacovelli.

Les politiques publiques financées par les crédits de cette mission visent donc, d'abord, à développer l'activité et la compétitivité des entreprises, dans un contexte de ralentissement de la croissance européenne. Ces politiques publiques concernent, en particulier, le développement international des entreprises et visent à élaborer un environnement conciliant, une concurrence saine entre acteurs économiques et la protection des consommateurs. Le premier objectif de cette mission est de favoriser l'adaptation de l'économie française aux nouveaux enjeux. Cette adaptation passera nécessairement par l'allégement des démarches administratives au travers de la mise en place d'une plateforme en ligne unique pour gérer les formalités de création, mais aussi par l'accès à l'innovation dans le cadre de la mission « French Tech » pour les start-up. Réguler, sécuriser et moderniser : tel est le second objectif de la mission que nous examinons aujourd'hui. La DGCCRF concentrera donc ses interventions sur les enquêtes au service de la lutte contre les fraudes économiques. C'est la condition pour protéger les entreprises, mais aussi les consommateurs. La DGCCRF devra prendre en compte les nouveaux modèles économiques et les risques émergents pour s'assurer de la loyauté des marchés. Le renforcement de l'efficacité des aides aux entreprises, l'amélioration de l'efficacité du soutien public à l'internationalisation des entreprises et la nécessité d'assurer le fonctionnement loyal et sécurisé des marchés sont autant d'enjeux auxquels il nous faut répondre. Tels sont les objectifs qui guident cette mission. Le déploiement de la 5G conduira l'Agence nationale des fréquences à jouer un rôle déterminant dans la régulation, la sécurisation et la modernisation de notre économie. Son action sera guidée par deux principes : confiance et transparence à l'égard des citoyens. Pour le programme 134, « Développement des entreprises et régulations », les autorisations d'engagement s'élèveront à 1 047,4 millions d'euros, contre 898,2 millions d'euros en 2019, soit une hausse de 15,1 %, et les crédits de paiement à 1047,4 millions d'euros, contre 912,3 millions d'euros l'an dernier, ce qui représente une hausse de 14,8 %. Au vu du temps qui m'est imparti, je souhaiterais revenir en particulier sur le programme 343, « Plan France Très haut débit Au-delà de l'enjeu économique et social de cette nouvelle économie numérique, le très haut débit permettra de désenclaver les territoires éloignés des grandes villes. Il s'agit là d'une demande forte de la part des élus locaux, que nous représentons dans cette assemblée et, à travers eux, de millions de Français. L'État a décidé un tel déploiement sur l'ensemble du territoire français d'ici à 2022 pour permettre à tous les citoyens d'accéder au numérique. Depuis la fin de l'année 2016, sous la présidence de François Hollande, 50 % de la population en bénéficie, avec un an d'avance sur le calendrier prévu. Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020, le programme prévoit la participation de l'État au financement de la couverture intégrale du territoire en internet fixe très haut débit, soit 3,3 milliards d'euros d'ici à 2022. Lancé en 2013, le plan France Très haut débit répond à un triple objectif : renforcer la compétitivité de notre économie et l'attractivité de la France ; développer les services publics innovants sur l'ensemble du territoire ; et, comme je l'ai rappelé, permettre l'accès au numérique pour tous les Français. Il est en effet urgent d'apporter une solution de connectivité aux foyers mal desservis. C'est pourquoi l'atteinte de cet objectif requiert l'utilisation de toutes les technologies. En prévoyant un guichet de la cohésion numérique, comme l'a annoncé le Premier ministre à Cahors le 14 décembre 2017, le plan France Très haut débit apporte une solution de connectivité aux foyers mal desservis. Une enveloppe de 100 millions d'euros attribuée pour proposer un soutien financier aux Français concernés pour l'installation d'équipements de réception d'internet. Le plan s'inscrit enfin dans l'ambition de long terme : doter le pays de nouvelles infrastructures de pointe, au travers de la généralisation de la couverture gigabit sur l'ensemble du territoire. Au total, l'État investira 3,3 milliards d'euros pour le déploiement du très haut débit. Le Gouvernement a rappelé l'exigence de tenir les objectifs, quitte à compléter les financements nécessaires pour que la France apparaisse en leader sur le déploiement du très haut débit. Nous ne pouvons que nous en féliciter. En 2020, les autorisations d'engagement du programme 343 s'élèveront à 330 millions d'euros et les crédits de paiement à 440 millions d'euros. Pour toutes les raisons évoquées, nous soutenons les crédits qui sont présentés. Ils constituent une réponse satisfaisante aux objectifs annoncés rendre plus efficaces les aides aux entreprises, renforcer leur compétitivité et permettre à tous les Français d'accéder aux mêmes ressources numériques sur l'ensemble du territoire. La parole

l'an dernier, pour un revenu moyen atteignant 5,8 millions d'euros. Cela va bien pour tous ceux qui ont perçu des dividendes records cette année, près de 51 milliards d'euros, et qui bénéficient en plus d'une allégée. Cela va bien pour les 100 premiers contribuables de France, qui, grâce à la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), ont gagné près de 1,7 million d'euros chacun sans pour autant investir dans l'économie réelle, comme le montre un rapport du Sénat. Vous nous dites que l'économie va mieux, que le niveau de chômage baisse et que l'emploi repart. C'est vrai, mais légèrement ... Vous oubliez de dire que ce qui a été créé est non pas de l'emploi, mais de l'activité. L'uberisation de la société crée de l'activité, mais pas de l'emploi. Dans votre vision de la société, nous aurons chacun un revenu, mais pas un salaire ni une protection sociale avec des droits rattachés. La réalité est que la part de personnes qui accédaient au marché du travail avec un CDD de moins d'un mois inférieure à 50 %. Elle est passée à plus de 70 % en 2019. Cela signifie que l'accès au monde du travail est marqué aujourd'hui par une très grande précarité. La réforme de l'allocation chômage que vous allez mettre en oeuvre touchera la moitié des personnes inscrites à Pôle emploi. De plus, 200 000 personnes n'auront plus accès à une indemnité. Ces gens disparaîtront des radars, mais ce sont des hommes et des femmes qui existeront toujours. Aujourd'hui, le marché du travail, ce sont des salariés pris en tenaille entre concurrence et rentabilité, au seul profit des actionnaires. ce n'est plus le marché du travail ; c'est le marché de la misère ! Que l'on songe à l'augmentation vertigineuse du nombre de travailleurs pauvres : plus d'un million de travailleurs vivent avec moins de 855 euros par mois. Voilà donc la réalité des chiffres Vous nous dites que l'économie va mieux. Oui, pour nos grands groupes. Mais la réalité est différente pour nos PME et TPE ! Vous dites que le coût du travail nuit à notre compétitivité. Mais le coût du capital, c'est-à-dire la charge des intérêts aux banques et les dividendes,

compétitivité et l'emploi (CICE) n'a été mis en place depuis la création et la transformation de ce dispositif, alors qu'il bénéficie pour plus de moitié aux très grands groupes. Les entreprises coûtent chaque année 200 milliards d'euros aux contribuables au travers de 6 000 dispositifs, de l'échelon local au niveau européen. Et vous refusez toujours de réorienter les aides fiscales en les destinant aux TPE-PME, qui en ont le plus besoin, ou, mieux, de les conditionner en contrepartie à des résultats en termes d'emploi, d'investissements ou de salaires. Alors, comment s'étonner des dérives ?

dont deux seulement ont été installées sur le site. Les six autres sont allées alimenter des sites roumains, polonais et espagnols appartenant au groupe ! En somme, le CICE aurait servi à développer des usines et donc des unités de production, voire peut-être des emplois, hors du territoire national, laissant des sites français fermer et des salariés être bientôt licenciés. Vous nous dites que l'économie va mieux et que tous les Français peuvent en être fiers. Tous Alors, pourquoi y a-t-il tant de colères chez les médecins et les personnels soignants, les enseignants, les facteurs, les forestiers de l'Office national des forêts (ONF), les pompiers, nos forces de sécurité, les agriculteurs, les étudiants, les cheminots, les retraités et les salariés du privé ? Peut-être parce que le taux de pauvreté augmente de 0,6 point en 2018, pour atteindre près de 15 % de la population. Peut-être parce que les inégalités se creusent comme jamais dans notre pays et que les salaires, dont le SMIC, que vous refusez d'augmenter, sont bloqués. Peut-être parce que, chaque jour, la solidarité se délite et le service public est sacrifié. Nous échangeons ici des chiffres, mais, en réalité, nous avons un débat profond avec vous. Pour vous, l'humain doit être sacrifié au nom de l'économie, de la croissance et de la réduction de la dette. Pour nous,

Il s'agit d'une mission au champ d'application très vaste et aux implications déterminantes pour le tissu économique de notre pays. Il y a lieu de se réjouir de la progression de ces crédits de paiement, puisqu'on constate une augmentation de 20 % entre 2019 et 2020. Mais l'essentiel de cette hausse de 2,3 milliards d'euros est lié au plan France Très haut débit et à la compensation carbone. Il s'agit de deux leviers déterminants pour faire évoluer notre économie vers un modèle à la fois plus ouvert sur le monde et moins polluant pour la planète. Mais cette transition ne doit, et ne pourra se réaliser qu'en associant dans un tel mouvement l'ensemble de nos entreprises. Je pense tout particulièrement à nos PME et entreprises de taille qui structurent l'économie de nos territoires. Elles doivent constituer la cible prioritaire de nos politiques publiques. Selon le sociologue Pierre Veltz, notre société, qui semble de plus en plus virtuelle, est en fait de plus en plus industrielle ; elle est même devenue hyper-industrielle. Pour que la France garde son rang dans la mondialisation, notre notre politique économique doit donc se doter d'une stratégie industrielle ambitieuse, fondée aussi bien sur l'innovation que sur la montée en gamme. La France doit donc amorcer sa reconquête industrielle en se dotant d'une stratégie ambitieuse et globale.

Les crédits de la mission « Économie » nous permettent d'avancer dans la direction que j'ai évoquée. Cependant, je partage le constat de notre excellent rapporteur Serge Babary : l'important volume de dépenses fiscales est encore trop peu tourné vers l'industrie. Le budget que nous examinons aujourd'hui comporte tout de même des avancées significatives. Cela vaut tout particulièrement pour l'effort fiscal réalisé pour la compétitivité des entreprises électro-intensives, qui se trouvent au coeur de notre tissu industriel.

cette mesure de responsabilité. Il s'agit de construire une fiscalité adaptée aux besoins spécifiques de ces acteurs indispensables à la chaîne de production industrielle. La logique reste la même : adapter notre fiscalité pour faciliter l'implantation de nos entreprises sur nos territoires. Le levier fiscal se révèle très puissant pour engager des transformations rapides. C'est ce qui explique l'accueil favorable que nous réservons au suramortissement pour nos PME ; le dispositif gagnera sans doute à être pérennisé. Il s'agit d'encourager nos entreprises à renouveler rapidement leur appareil productif, afin qu'elles demeurent compétitives sur les marchés internationaux. Bien entendu, l'industrie ne saurait constituer l'alpha et l'oméga de notre politique économique. D'autres acteurs contribuent aussi au dynamisme économique dans nos territoires. Je pense notamment à l'artisanat et au commerce de proximité. À ce titre, je soutiens

Mes chers collègues, je crois que notre commission a largement contribué à l'amélioration de l'utilisation des crédits prévus par cette mission. Dorénavant, nos efforts devront nous conduire à réduire les impôts de production, qui grèvent la compétitivité des entreprises implantées sur notre territoire, mais permettent d'importantes recettes pour les collectivités, déjà fort sollicitées. C'est donc dans le cadre d'une réforme plus large de la fiscalité locale qu'il faudra s'y attaquer en intégrant l'autonomie fiscale de nos collectivités. Le défi est donc essentiel pour améliorer la compétitivité de notre pays tout en soutenant l'activité dans nos territoires. Nous vous encourageons dans cette action. La

améliorées. Si une hausse apparente des crédits d'environ 6 % nous est présentée aujourd'hui, elle est principalement liée à la compensation carbone pour les entreprises électro-intensives. C'est ainsi une augmentation de budget en trompe-l'oeil qui est proposée. La logique de baisse des dépenses publiques et de désengagement est aussi à l'oeuvre ici. L'on peut s'en inquiéter, tant notre pays aurait besoin de soutenir son économie, notamment pour revitaliser les territoires ruraux, mais aussi pour accompagner accompagner la nécessaire transition écologique des entreprises. Ainsi, les dispositifs à destination des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, qui devraient représenter le coeur de cette mission, sont en diminution depuis plusieurs années. Je déplore donc, comme nombre de mes collègues, la diminution des crédits du Fisac, placé en gestion extinctive depuis cette année. justifie cette disparition en mettant en avant le programme Action coeur de ville. Si celui-ci est intéressant, il ne concerne que 222 villes et n'a donc pas la même cible que le Fisac, lequel s'adresse avant tout aux petites communes. Ayant été maire d'une commune semi-rurale touchée par des difficultés de maintien des petits commerces, je suis très attaché à ce dispositif de soutien à l'économie de proximité,

Toujours sur la question de la mise à mal des dispositifs de soutien à l'économie de proximité, notamment en zone rurale, je regrette la baisse des financements des chambres de commerce et de l'industrie. elles ont perdu 28 % de leurs emplois alors que leur rôle est important sur les territoires, notamment pour l'accompagnement de proximité.

et PME, qui ont, rappelons-le, des difficultés à accéder au crédit bancaire. De plus, comme le précise le rapport, Bpifrance étudie la possibilité de mettre en place un prêt sans garantie qui financerait les investissements des PME et ETI afin de réduire leur empreinte énergétique, dispositif qui ne pourrait pas voir le jour sans sécurisation de l'activité de garantie. Je soutiendrai donc les amendements de la commission visant à abonder ce dispositif. Je souhaite également aborder les moyens de la DGCCRF. Certes, ses effectifs sont conservés pour 2020. On pourrait déjà s'en satisfaire, puisque la tendance est plutôt à la baisse dans les administrations. Mais, malgré tout, son budget est passé d'environ 242 millions d'euros à 226 millions d'euros depuis 2018. Cela constitue une baisse significative et amène à s'interroger sur sa capacité à effectuer les contrôles nécessaires, à l'heure où interviennent des scandales sanitaires qui inquiètent à juste titre nos concitoyens. Pour prendre l'exemple du secteur agricole, la signature du CETA, souhaitée par le Gouvernement, devrait l'amener à renforcer les moyens de contrôle, au lieu de simplement stabiliser les effectifs. Si l'on peut encore espérer que la France ne ratifiera pas ce traité, il convient de manière générale de protéger les agriculteurs des concurrences déloyales qu'ils subissent l'importation de produits ne respectant pas les normes européennes. Le plan France Très haut débit est marqué par une hausse des décaissements. Il est ici important de soutenir une couverture du territoire en réseau numérique, notamment pour les territoires ruraux, qui peuvent souffrir d'un défaut d'attractivité faute d'accès à des réseaux satisfaisants.

Elle illustre finalement et malheureusement très bien les risques du « en même temps ». Elle fait en effet passer nos avis de favorables à défavorables selon l'angle d'observation. On passe du positif quand on regarde l'augmentation de près de 20 % des crédits de la mission par rapport à 2019, au négatif quand on constate l'absence de véritable stratégie industrielle. On passe de l'enthousiasme quand on se félicite des engagements sur le plan France Très haut débit, à la déception quand on réalise que c'est au détriment du Fisac, dont l'extinction est proche. Or une politique économique et industrielle ne peut se mener que si elle a deux orientations majeures : d'une part, une vision stratégique nationale et européenne qui fixe un cap ; d'autre part, une ambition et des outils performants qui irriguent le territoire. C'est l'absence d'articulation entre ces deux axes qui nous semble constituer un manque. Comme la plupart des pays développés, la France a été confrontée à la désindustrialisation de son économie, la part de l'industrie dans le produit intérieur brut étant passée de 24 % en 1980 à 12,6 % en 2016. Ainsi, 25 % des emplois industriels ont disparu depuis l'an 2000. Une telle situation peut être corrigée à condition que l'État se donne les moyens d'accompagner efficacement son industrie et les territoires, se comporte en véritable stratège. Malheureusement, nous observons aujourd'hui un comportement relevant plus de l'État pompier que de l'État stratège. C'est ce que constate et dénonce notamment notre collègue Valérie Létard dans son rapport d'information sur les enjeux de la filière sidérurgique dans la France du XXI siècle. Qui pilote la stratégie au sein du Gouvernement ? Y a-t-il un ministre qui ne soit pas juste le sauveteur des plans de licenciements ? Il y a nécessité et urgence de tracer un plan stratégique pour créer de l'emploi, pour retrouver une place majeure dans l'industrie mondiale, pour s'adapter à l'économie du numérique et climatique et pour inciter à la recherche dans ces domaines.

Il faut ensuite diffuser et irriguer notre territoire avec les bons outils et les bonnes infrastructures. Je souhaite aborder, d'une part, le numérique et, d'autre part, l'artisanat et le commerce local.

C'était attendu par les entreprises, par les collectivités locales, qui ont pris toute leur part dans le déploiement des infrastructures, en particulier en milieu rural, et, bien évidemment, Je soutiens les propositions de Mme la rapporteure pour avis Anne-Catherine Loisier, qui souhaite rendre possible l'équipement des vingt-sept départements et de toutes les zones rurales en attente, afin de « booster » notre économie.

Or nous pouvons tous ici témoigner de l'utilité et de l'intérêt de ce fonds pour maintenir l'artisanat et le commerce, en particulier dans les zones rurales. Le de sauver de l'activité économique de proximité, de conserver une vie et une attractivité dans les communes rurales et dans les centres-bourgs de centaines de petites communes qui ne sont pas incluses dans les opérations de

d'un sujet auquel je suis très sensible en tant que membre de la commission des affaires économiques et de la délégation sénatoriale aux entreprises. Mais c'est surtout la représentante d'un territoire rural et de montagne qui s'exprime devant vous aujourd'hui, car l'économie des territoires est abandonnée par l'État. Bien entendu, sur le papier, l'économie relève désormais de la compétence des régions. Mais, dans nos communes, dans nos vallées et dans nos campagnes, l'artisanat et les petits commerces sont à la peine, car les régions aident prioritairement des secteurs d'activité stratégiques. Qui d'autre que l'État peut être garant d'une équité territoriale ? Selon que vous habitez dans telle ou telle commune, selon que vous êtes en Auvergne-Rhône-Alpes ou en région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous n'aurez pas les mêmes aides et vous ne bénéficierez pas du même dispositif d'accompagnement. C'est pourquoi il est important que l'État ne se désengage pas de l'économie des territoires au profit des seules régions. les collectivités « XXL », qui sont plus préoccupées par les métropoles et par les grandes agglomérations et qui doivent être plus attractives pour les investisseurs et plus compétitives pour rivaliser, notamment, avec leurs voisines européennes.

Je voudrais également dénoncer la baisse significative des crédits alloués aux métiers d'art. Alors que nous devons reconstruire Notre-Dame de Paris et qu'une souscription nationale a été lancée, la dotation budgétaire de l'Institut national Cette incohérence entre les annonces et les actes doit être soulignée et corrigée. En effet, au-delà d'un patrimoine immatériel faisant partie de notre culture, les 281 métiers recensés actuellement doivent être encouragés et tout doit être mis en oeuvre pour qu'ils puissent recruter de nouveaux talents. Alors que nous avons besoin des savoir-faire et de l'excellence française dans de nombreux domaines d'activité, il n'est pas envisageable de faire des économies au détriment des métiers d'art.

loi Pacte, a entraîné une transformation du modèle économique des CCI consistant désormais à déployer une démarche commerciale. Mais la baisse de financement ne pourra être que partiellement compensée par le développement de prestations tarifées. En effet, les entreprises ayant besoin d'un accompagnement ne pouvant pas s'offrir des prestations trop onéreuses, les CCI ne pourront donc proposer que des tarifs peu élevés. Ceux-ci seront insuffisants pour compenser la baisse de taxe Dans ce contexte, alors que les TPE et PME sont redevables de la TFC, elles devront désormais payer pour des services qui étaient auparavant gratuits. Certaines entreprises se retrouveront même en concurrence avec les CCI sur des secteurs d'activité, alors qu'elles financent ces CCI par la TFC et que ces dernières pourront proposer des prix plus avantageux. Le réseau ne pourra donc plus remplir ses missions de service public de proximité complet et permanent, rôle essentiel pour le tissu économique local.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette mission a pour objectif de soutenir les dynamiques économiques du pays et, par voie de conséquence, les dynamiques économiques et sociales des territoires. De manière globale, sur l'ensemble de la mission, on ne peut que déplorer la baisse du plafond d'emplois, 294 équivalents temps plein étant retirés. Cette baisse de ressources humaines s'inscrit finalement dans la continuité de la politique du Gouvernement, qui vise à réduire le service public. Il faut s'attacher à regarder les conséquences de ces choix politiques sur l'économie de nos territoires, notamment sur celle de la ruralité. Pour cela, il nous paraît primordial d'étudier les choix faits sur le Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce sur les chambres de commerce et d'industrie et sur le plan France Très haut débit. Le Programme 134, « Développement des entreprises et régulations », cristallise sensiblement les conséquences des choix budgétaires du Gouvernement en zone rurale.

Après avoir subi plusieurs années de baisse de son budget, le Fisac se retrouve désormais fondu dans l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Si cette réforme répond à un besoin des collectivités, elle ne leur apporte aucune plus-value financière. En effet, cette nouvelle agence correspond uniquement à une mise en commun de moyens, et non à une politique de redynamisation ambitieuse qui permettrait de valoriser nos territoires, ainsi que les femmes et les hommes qui y travaillent et y vivent. Finalement, le Gouvernement choisit d'abandonner un dispositif qui fonctionnait bien, démontrant qu'il délaisse nos régions, nos artisans et nos commerçants. Il en est de même pour les chambres de commerce et d'industrie. En effet, la mise en place de la loi Pacte, qui devait, selon le ministre de l'économie, « transformer profondément les chambres de commerce et d'industrie », a surtout entraîné une chute de leurs ressources fiscales. En fragilisant les CCI, ces piliers solides sur lesquels nos régions pouvaient s'appuyer, on fragilise l'ensemble du tissu économique. L'État choisit de se retirer inexorablement des politiques économiques de proximité et de laisser peser les dépenses sur les autres collectivités. Pourtant, nos chambres les plus vulnérables se situent en zone rurale. Ces choix budgétaires sont étonnants, car les CCI assurent un rôle important de formation, de diffusion de l'information et de prévention auprès des TPE et PME. Ce sont des institutions vers lesquelles les entrepreneurs, les commerçants et les artisans peuvent se tourner pour être accompagnés et conseillés efficacement dans leurs démarches.

et environnementales des territoires. Leur rôle est d'autant plus important dans les zones rurales. Elles connaissent bien ces hommes et ces femmes qui oeuvrent à animer la vie de nos départements ruraux. Ce sont aussi elles qui tissent et entretiennent le maillage territorial, donc animent la vie économique et sociale des départements. et républicain regrette que l'amendement visant à garantir un plancher de financement, qui aurait pu assurer le maintien des CCI fragilisées, n'ait pas été intégré dans le projet de loi de finances pour 2020. Madame la secrétaire d'État, au moment de la loi Pacte, vous aviez évoqué une aide pour les structures fragiles, ainsi qu'une nouvelle péréquation en faveur des CCI rurales. Aujourd'hui, une fois de plus, en présentant ce budget, vous ne tenez pas vos promesses. À travers les CCI, c'est l'ensemble du tissu économique des territoires que vous mettez en péril, des territoires qui subissent une dévitalisation et un éloignement accentués par la fracture numérique. Cela nous amène à notre dernier point : le plan France Très haut débit. On pourrait penser que, avec la hausse des crédits de paiement, le budget alloué à ce plan serait en forte hausse. Malheureusement, cette augmentation ne résulte que des mouvements comptables des années précédentes. L'investissement dans les réseaux d'initiative publique (RIP) avait été évalué à environ 14 milliards d'euros. L'État s'était engagé à hauteur de 3,3 milliards d'euros d'ici à 2022, soit la moitié du financement public. Nous souhaitons vous rappeler l'importance de l'accès au numérique pour les TPE et les PME des territoires ruraux. Ces entreprises ont besoin de ne pas être tenues à l'écart des outils numériques. Il en va de leur efficacité et de leur compétitivité comme de leur développement. Or, si les opérateurs téléphoniques et l'État préparent actuellement l'arrivée de la 5G, près de 15 % du territoire national n'a toujours pas accès au très haut débit. Eh oui ! Même si nous nous félicitons de leur mise en oeuvre, les crédits de paiement alloués à cette mission ne sont pas suffisants pour permettre aux 2 600 communes en zones blanches ou grises d'avoir accès au très haut débit d'ici à 2022. Cette enveloppe ne fera progresser que de 2 % le taux de couverture très haut débit, le faisant passer de 83 % en 2019 à 85 % en 2020. n'est donc pas du tout à la hauteur des objectifs annoncés par le Gouvernement d'ici à la fin du quinquennat. De plus, nous vous rappelons que si le développement de la 5G doit être soutenu, il ne doit pas se faire au détriment de l'arrivée de la 4G dans les territoires ruraux. Le numérique doit être accessible à tous. Pour conclure, le budget global de cette mission ne répond pas aux réels besoins de développement économique de tous nos territoires. Nous le regrettons, car il risque d'accentuer les inégalités entre ruraux et urbains, tout en délaissant des dispositifs et des institutions qui ont pourtant fait la preuve de leur efficacité. La parole

En 2004, notre ancien collègue, Philippe Leroy, disparu cet été, s'était battu avec force pour que les collectivités aient le droit d'intervenir pour aménager numériquement leur territoire. L'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, texte fondateur de l'aménagement numérique du territoire, avait été acquis de haute lutte. Par la suite, et jusqu'à fin 2017, non seulement l'intervention publique s'est retrouvée de moins en moins contestée, mais surtout son opportunité et sa nécessité absolue n'ont jamais été démenties, comme en témoigne le fort soutien de l'État au travers du plan France Très haut débit en 2013. les réseaux d'initiative publique déploient massivement des prises pourtant trois fois plus longues et complexes à construire que celles de la zone d'initiative privée. Il faut les mêmes ressources humaines, techniques et financières pour déployer une prise en zone publique que trois prises en zone privée.

Comment soutenir que les 140 millions d'euros disponibles pour le guichet 2.0 suffiront, alors qu'il reste un peu plus de 3 millions de foyers à fibrer sur 27 départements, ce qui nécessite environ 600 millions d'euros d'accompagnement de l'État ? Selon notre estimation, l'ensemble des dossiers prêts à être déposés dès réouverture du guichet représentent près de 462 millions d'euros de demande de Fonds Le seul dossier breton nécessite pour ses quatre départements 200 millions d'euros. La régie Auvergne numérique escompte, pour ses quatre départements, un peu plus de 100 millions d'euros. En outre, il reste une douzaine d'autres départements prêts à déposer une demande de FSN Pas besoin d'avoir fait l'ENA ou Polytechnique pour comprendre que le compte n'y est pas et que les parlementaires doivent achever le travail dans le cadre de ce projet de loi de finances. Je me félicite d'ailleurs des nombreuses initiatives transpartisanes, comme des interventions à cette tribune,

Pour valider son propos selon lequel le budget actuel du plan France Très haut débit suffira pour atteindre les 100 % FTTH (), le Gouvernement prévoirait d'aider les derniers territoires de manière particulièrement minimaliste, alors même que les 75 premiers départements à être partis sur le 100 % FTTH ont été massivement aidés par l'État, celui-ci étant même parfois le premier cofinanceur des RIP. Le comble, c'est que le reste à faire est bien plus coûteux que ce qui a déjà été réalisé. Pour illustrer mon propos, à régime d'aide inchangé, la régie Auvergne numérique ne pourrait pas financer le 100 % FTTH et devrait se limiter. C'est donc l'inverse que l'État aurait dû faire ! Pour achever cet assaut d'iniquités entre les départements français, il est question pour l'État d'accompagner uniquement le déploiement jusqu'à 92 % des logements, avec le mythe tenace chez certains décideurs hors sol qu'il ne faut pas financer le fibrage des gîtes de haute montagne. Comme si nous avions en France 8 % de gîtes de haute montagne

Le plan France Très haut débit est une réussite exceptionnelle. Ne laissons pas quelques acteurs hors sol, déconnectés des réalités de nos territoires et des attentes de nos concitoyens, décider seuls de ce qui est bon pour eux. Votons les crédits nécessaires pour assurer une égalité des Français devant l'accès à internet, et une égalité des territoires dans l'accompagnement de la puissance publique. Très bien

Les résultats de notre politique sont perceptibles. Dans un contexte international tendu, marqué par la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis et par les incertitudes politiques en Europe, la contribution du commerce extérieur à la croissance du pays est redevenue positive et la France est désormais un territoire très attractif au sein de la zone euro pour les investissements Je rappelle que nous sommes en première position pour l'attraction des investissements industriels, grâce à une politique d'attractivité, et pour les investissements en R&D. La croissance est solide : 1,4 % en 2019 et 1,3 % prévu pour l'année prochaine. Les résultats de l'Insee montrent que nous sommes toujours dans cette trajectoire, trimestre après trimestre. L'investissement des entreprises est reparti à la hausse, en progression de 7 milliards d'euros en deux ans, un montant trois fois supérieur à la progression annuelle moyenne des investissements entre 2012 et 2016. Le niveau de chômage, qui a

beaucoup plus des emplois à durée indéterminée et des emplois durables que dans le passé. Nous avons recréé des emplois industriels, ce qui n'était pas arrivé depuis 2000. Ce sont des faits, bien loin de certaines caricatures.

visant à réduire le nombre de contrats courts, car c'est bien une réalité inadmissible. Parlons-en ! Avec ce budget 2020, nous poursuivons cette politique. Notre premier objectif est bien de soutenir les entreprises françaises, notamment les entreprises industrielles, en améliorant leur compétitivité. Je rappelle que les impôts baisseront de 1 milliard d'euros en 2020 pour nos entreprises et de 13 milliards d'euros sur l'ensemble du quinquennat. La trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés, initiée par la loi de finances pour 2018, est poursuivie en 2020, avec pour cible, conformément à l'engagement du Gouvernement,

Dans le prolongement de ces réformes, nous souhaitons, d'ici au projet de loi de finances pour 2021, travailler sur l'allégement des impôts de production. Ceux-ci représentent 70 milliards d'euros. Ils sont trois fois plus élevés en montant que ceux de l'Allemagne, sept fois plus en pourcentage du PIB.

d'autres possibilités existent. J'entends des régions et des collectivités locales qui veulent participer à la trajectoire de baisse des impôts de production ; nous serons évidemment à l'écoute de ces demandes. Outre ces allégements d'impôts, nous continuons d'assurer un soutien

à la « compensation carbone ». Ce dispositif, qui permet de compenser le coût des quotas carbone pour les industriels électro-intensifs, vise à accompagner l'adaptation des équipements des entreprises et à protéger les entreprises industrielles concernées

un effort significatif, tout en accompagnant ces industriels dans une meilleure maîtrise de leur utilisation de l'énergie. Je veux aussi rassurer beaucoup d'entre vous

Enfin, la taille des fonds de garantie au bilan de Bpifrance Financement montre qu'il n'y a aucun désinvestissement de la part de l'État dans le pilotage de ces fonds. Les octrois de garantie devraient d'ailleurs légèrement augmenter en 2019 par rapport à 2018, sans que la solvabilité de Bpifrance Financement en soit réellement affectée. De manière générale, sur la politique industrielle, 31 % des concours de Bpifrance sont consacrés aux entreprises industrielles, alors qu'elles ne représentent qu'à peine plus de 10

Nous soutenons, enfin, la compétitivité des entreprises à l'export. C'est la vocation de la réforme du service public de l'export mise en oeuvre par Business France, qui regroupe au sein de la l'ensemble des acteurs publics et privés pour offrir aux entreprises un accompagnement plus efficient, en phase avec leurs besoins. Le Le démarrage de ce projet est très satisfaisant. Le soutien que nous assurons aux entreprises est plus particulièrement orienté vers l'innovation, la politique du Gouvernement en la matière s'inscrivant dans un cadre rénové. Des mesures de simplification et de rationalisation ont déjà été prises depuis plusieurs années, instituant Bpifrance comme guichet unique pour la grande majorité des dispositifs de soutien à l'innovation. En outre, le Fonds pour l'innovation et l'industrie est désormais pleinement opérationnel. Par

5 millions de prises équivalentes avaient été déployées. Soyons capables de saluer cet effort majeur du Gouvernement, qui a permis de rattraper une partie de notre retard. En 2020, nous livrerons l'objectif de couverture en bon débit, soit 8 mégabits

des grands pays d'Europe, si l'on compare avec le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Notre action, qui montre son efficacité, se poursuit dans chaque territoire. Nous faisons évoluer nos modalités d'action dans les territoires, ce qui a conduit, depuis 2017, à prévoir une extinction progressive de dispositifs traditionnels comme le Fisac. Toutefois, ces dispositifs sont remplacés. Le Gouvernement a fait le choix, qu'il assume, de renouveler complètement sa façon d'opérer, à travers la mise en place de l'Agence nationale

Par ailleurs, je vous rappelle le lancement d'une stratégie nationale pour l'artisanat et le commerce de proximité, destinée spécifiquement aux TPE et PME.

mais, si l'on veut respecter le nouvel objectif de généralisation de la fibre jusqu'à l'abonné d'ici à 2025, il est impératif d'ouvrir dès 2020 de nouvelles autorisations d'engagement à hauteur de 322 millions d'euros. Sans cela, même avec un nouveau cahier des charges plus restrictif et des marchés resserrés, toutes les collectivités ne pourront pas lancer leurs projets et être au rendez-vous de 2025.

émet également un avis défavorable. Tout d'abord, nous avons tenu notre engagement de rouvrir le guichet, comme je l'avais indiqué ici même l'an dernier. Ensuite, nous n'avons pas besoin, dès 2020,

avis. Plus de 60 000 entreprises, dont 90 % sont des TPE, bénéficient chaque année de prêts garantis par Bpifrance pour un montant total d'environ 8,7 milliards d'euros. d'euros. Cette garantie comble une faille du marché et assure l'accès au crédit de toutes les entreprises, y compris celles qui sont les plus fragiles et les plus exposées à la concurrence. Depuis deux ans, le Gouvernement entend assécher complètement le financement de l'activité de garantie de Bpifrance par dotation budgétaire, alors que l'établissement s'appuyait les années précédentes sur une dotation qui oscillait entre 20 et 40 millions d'euros. La suppression de cette dotation budgétaire signerait dès 2021 l'arrêt de mort des activités de garantie. Madame la secrétaire d'État, je vous assure que, malheureusement,

nous paraît donc incohérent. C'est pourquoi cet amendement tend non seulement à rétablir le Fisac, mais aussi à porter sa dotation à 36 millions d'euros. Il n'est tout simplement pas possible de mener des politiques crédibles avec des montants plus modestes. Les trois

et la gouvernance des pôles de compétitivité qui permettent à l'État de cofinancer avec les régions le fonctionnement de ces pôles. Le rôle de ces pôles est en effet essentiel. La baisse des crédits est incohérente avec les objectifs du Gouvernement en matière de développement industriel et d'innovation annoncés dans le pacte productif.

la commission ? Le programme 134 concentrera, à partir de 2020, l'ensemble des crédits affectés aux pôles de compétitivité. Cependant, ces crédits sont largement insuffisants pour permettre une véritable dynamique à même de renforcer l'attractivité des pôles existants. Par ailleurs, ces crédits ont vocation à baisser progressivement au cours des prochaines années, puisqu'il faudra laisser la place aux régions qui disposent de la compétence de développement économique. C'est pourquoi la commission demande l'avis du Gouvernement

au soutien et à la promotion des métiers d'art afin qu'ils atteignent 2,25 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. Ces crédits financeront essentiellement l'action de l'Institut national des métiers d'art (INMA) et de l'Institut supérieur des métiers (ISM). Le projet de loi de finances pour 2020 ne prévoit en effet aucun crédit pour ces instituts, alors que 2,25 millions d'euros étaient inscrits en loi de finances initiale pour 2019.

D'après les informations qui nous ont été transmises, la disparition de la dotation budgétaire sur le programme 134 ne devrait pas remettre en cause le financement de l'agence en 2020. Toutefois, comme nous souhaitons être rassurés sur ce point, nous demandons l'avis du Gouvernement.

engagées en faveur de l'amélioration de la performance environnementale et de leur outil de production les moyens de faire face au mur d'investissements auquel elles sont confrontées.

en restructuration rencontrant des difficultés à accéder au marché du crédit, le fonds pour le développement économique et social (FDES). L'intervention de l'État en faveur d'entreprises structurellement viables, mais confrontées à des difficultés temporaires d'accès au crédit, est indispensable pour certains secteurs d'activités en difficulté et pour certains territoires particulièrement touchés par la désindustrialisation.

fort effet de levier sur les financements privés, de même qu'une dynamique collective vertueuse. C'est précisément la raison d'être de cet amendement, qui s'appuie sur la capacité d'intervention substantielle de l'État en la matière. Cette mesure ne ne mettra pas en péril les finances de l'État : elle montrera juste que celui-ci est au rendez-vous pour accompagner les projets industriels. Quel est l'avis de la commission ?

Compte tenu du caractère mécanique de ces dépenses, les crédits de cette mission sont évaluatifs, c'est-à-dire qu'ils ne constituent pas un plafond, à la différence des crédits des autres missions budgétaires. La mission est composée de deux programmes, l'un consacré aux remboursements et dégrèvements d'impôts d'État, l'autre aux remboursements et dégrèvements d'impôts directs locaux. Pour 2020, 141 milliards d'euros de crédits sont demandés au titre de la présente mission, en augmentation de 5 milliards d'euros par rapport à la loi de finances pour 2019. L'augmentation des impôts d'État s'explique notamment par la mise en oeuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, mais également par la hausse des restitutions de TVA et d'importants contentieux fiscaux. hausse des impôts locaux s'explique principalement par le coût croissant du dégrèvement de la taxe d'habitation en faveur de 80 % des ménages. Pour 2020, les remboursements et dégrèvements d'impôts d'État sont évalués à 118 milliards d'euros, en augmentation de près de 2 milliards d'euros par rapport à 2019. Leur hausse est quasi ininterrompue depuis 2010. D'abord, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) continue de peser sur la mission. Le coût prévu du dispositif pour 2020 est cependant en forte baisse. Alors qu'il atteignait presque 20 milliards d'euros en 2019, la prévision pour 2020 est de 9 milliards d'euros.

pour renforcer la lutte contre la fraude fiscale. Pour cela, l'information doit être décloisonnée et les services doivent travailler de façon coordonnée, aux échelons tant national qu'européen et international. Je considère en outre que les moyens humains doivent être renforcés et mieux spécialisés.

publiques afin de mieux répartir la charge de la TVA en révisant les taux d'imposition des produits et des services de première nécessité qui contribuent au maintien de la dignité des personnes. Nous avons déjà eu ce débat dans l'hémicycle. Je sais que les taux réduits font l'objet d'un encadrement strict par le droit de C'est pourquoi je demande que la France défende l'extension des taux réduits et super-réduits à l'échelon européen. En 2015, une initiative sénatoriale transpartisane a permis de réduire à 5,5 % le taux de TVA applicable aux protections hygiéniques féminines. Il faut poursuivre l'extension de ce taux réduit ; le Sénat l'a fait pour les protections hygiéniques pour les personnes âgées, mais l'Assemblée nationale s'y est opposée, au motif que c'était contraire au droit européen.

À titre personnel, je fais plutôt partie des sceptiques. J'observe que notre encours de dette négociable non seulement ne faiblit pas, mais devrait encore augmenter de 4,5 %. La dette publique devrait prospérer atteindre 98,7 % du PIB à la fin de l'année. Nous continuons ainsi à imposer à nos enfants une charge considérable et nous ne savons même pas s'ils pourront un jour la rembourser. Le poids de la dette nous éloigne encore un peu plus de nos partenaires européens.

On nous accuse souvent de jouer les Cassandre en alertant sur le risque d'une remontée des taux qui ne s'est pas matérialisée et qui a de grandes chances de ne pas se concrétiser ces prochaines années. Pour autant,

sur un réveil qui pourrait être douloureux. Notre collègue Philippe Dallier avait proposé à la commission des finances d'élaborer des scenarii de remontée des taux, de façon à pouvoir alerter

même si elle était infime -soit soutenable pour nos finances publiques, d'autant que nous venons d'apprendre la reprise de la dette hospitalière.

En 2018, plus du quart des dépenses de ce compte n'avaient aucun lien avec l'État actionnaire. En second lieu, la capacité d'action du Parlement est foulée aux pieds par la confidentialité des opérations de cessions.

Des propositions existent pour définir un meilleur équilibre des pouvoirs dans l'examen de ce compte. J'ai moi-même eu l'occasion d'en formuler l'an dernier. Ces réserves préliminaires exposées, j'en viens à la présentation des crédits de ce

Paris, en revanche, le Gouvernement se fait plus discret sur le processus de recueil des soutiens à la proposition de loi déposée en application de l'article 11 de la Constitution. Engagé le 13 juin dernier, ce processus doit se poursuivre jusqu'à la mi-mars 2020, le projet de cession étant entre-temps suspendu. Le Sénat a exprimé son opposition à ces deux cessions. Au-delà des débats relatifs au caractère stratégique de ces actifs, laissez-moi vous faire part des conséquences budgétaires Les dividendes seront perdus, à hauteur d'environ 200 millions d'euros chaque année. Voilà qui renforcera une tendance de fond : entre 2012 et 2019, les dividendes perçus par l'État ont été divisés par deux. Surtout, ces cessions réduiront fortement les marges de manoeuvre de l'État actionnaire. Depuis son entrée en fonction, le Gouvernement a asséché de 60 % le solde de ce L'exécutif semble avoir oublié que le b.a.-ba de tout gestionnaire d'actif est la diversification de son portefeuille. Pour qualifier sa stratégie, le Gouvernement convoque un élément de langage : il parle de « respiration » du portefeuille. Pardonnez ma brutalité, mais j'y vois plutôt le dernier souffle de l'État actionnaire ! Pourtant, les défis à relever sont nombreux et cruciaux pour l'avenir de notre pays : je pense en particulier à la transition énergétique et à ses conséquences pour EDF. De ce point de vue, je ne peux cautionner le choix qu'a fait le Gouvernement de mobiliser ce compte pour le désendettement de l'État. Le symbole ne doit pas s'opérer à rebours des intérêts patrimoniaux de l'État, alors que les conditions de marché sont exceptionnelles. Permettez-moi de citer un ancien ministre, qui indiquait en 2016 devant la commission des finances que « patrimonialement, ce serait se tirer une balle dans le pied que d'utiliser le capital du compte d'affectation Entre-temps, l'ancien ministre a quitté Bercy pour l'Élysée et son regard semble avoir changé, alors que le contexte macroéconomique demeure similaire. Quel est le risque ? C'est que ce compte en faisant fi des considérations patrimoniales. La dette publique tutoie désormais le seuil hautement symbolique des 100 % du PIB. La contribution au désendettement prévue explique à elle seule le reflux de 0,1 point de PIB du ratio qu'escompte le Gouvernement en 2020.

mes chers collègues, que je ne saurais vous éclairer sur ce point. En revanche, je suis en mesure de vous faire part de l'usine à gaz budgétaire que met en oeuvre le Gouvernement. Excellent est volontiers moderniste : on convoque nombre d'anglicismes pour étayer ce qui reste une opération de débudgétisation, qui s'effectue au détriment des capacités d'analyse du Parlement.

Son actualisation est prévue à l'échéance pour le moins opportune du 1 janvier 2023. La révision éventuelle serait effectuée à la fois pour l'avenir et pour le passé : le trop versé pourrait être répercuté sur la rémunération ultérieure.

monsieur le ministre, mes chers collègues, je me fais le porte-parole de Jean Bizet, qui a pris ma suite comme rapporteur spécial pour les crédits de la mission « Investissements d'avenir ». Je suis heureuse de constater que les crédits demandés pour 2020 s'élèvent à 2 milliards d'euros, soit près du double du montant qui a été voté l'année dernière. Cela témoigne incontestablement d'investissements d'avenir, le PIA 3. La nouvelle programmation triennale prévoit ensuite une stabilisation autour de 2 milliards d'euros en 2021 et 2022. Au-delà de cette augmentation des crédits, nous pouvons affirmer qu'après un démarrage relativement poussif le PIA 3 est désormais pleinement mis en oeuvre. Quatre chiffres en témoignent : 90 % des autorisations sont consommées, 26 conventions État-opérateurs ont été signées sur 27, 820 projets sont aujourd'hui en phase active, donnant lieu à un investissement de 1,7

cette ambition. Nous nous félicitons que figure le chantier de l'intelligence artificielle. L'Europe et la France ont accumulé trop de retard dans ce domaine ; le concours de 75 millions d'euros apporté par le PIA 3 à la constitution des nouveaux instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle (3IA) n'est donc pas de trop. Une certaine dispersion- pour ne pas dire un saupoudrage -des fonds publics en faveur de l'intelligence artificielle peut toutefois être déplorée. Nous sommes plus dubitatifs quant à la thématique « Recherche dans le domaine du sport de très haute performance », qui se voit dotée de 20 millions d'euros au sein de cette même parfaitement intégré aux objectifs du PIA. Il en va de même, cette fois dans le domaine culturel, du projet, repoussé mais pas enterré, de financer la rénovation du Grand Palais par les crédits du PIA. La commission des finances est vivement opposée à ce type de détournements. Il ne s'agit pas de remettre en cause le bien-fondé d'un soutien public à de telles initiatives ; nous constatons simplement que les actions du PIA 3 ne constituent pas l'instrument adapté. les PIA ont été instaurés de manière à accroître le potentiel de croissance de l'économie française en investissant dans des chantiers prioritaires définis par un État stratège, et non pour concourir au financement d'événements ponctuels ou à la rénovation de notre patrimoine. L'année 2020 marquera le dixième anniversaire du premier PIA ; il est donc l'heure d'en tirer un premier bilan. Celui-ci nécessite une évaluation minutieuse et complexe. En 2010, le PIA 1 avait été présenté comme une initiative exceptionnelle, un grand emprunt visant à investir dans l'avenir et à tourner la page de la crise. Dix ans et deux PIA plus tard, on pourrait craindre une certaine forme de banalisation de l'exceptionnel. Le secrétariat général pour l'investissement, ainsi que les opérateurs, tendent au contraire à considérer que c'est précisément cette stabilité qui fait la force du dispositif : elle contribue à faire du label PIA un repère que les agents économiques se sont approprié et qui tend à apporter de la crédibilité au soutien public à l'innovation de long terme. C'est ce débat qu'il faudra trancher. En l'état, la commission vous propose d'adopter sans modification les crédits de cette mission. Très bien

opère actuellement un recentrage de son portefeuille sur un nombre très réduit d'actifs : EDF représente aujourd'hui la moitié de la valeur de son portefeuille. Or cela prive l'État de marges de manoeuvre dans le cas où des liquidités pour protéger une entreprise fragile ou menacée. Surtout, le fameux fonds pour l'innovation et l'industrie, qui est alimenté par le produit des cessions et doit générer un rendement de 250 millions d'euros

plus stable que ne le permettrait un financement par les dividendes. Or il est maintenant prévu pour 2023 une clause de revoyure qui permettra de diminuer le rendement de ce fonds s'il se révèle supérieur à celui du marché, ce qui est plutôt de bonne gestion, mais ne manquera pas d'arriver. Même la stabilité du financement n'est donc à ce jour plus garantie.

Mes chers collègues, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque unité de discussion comprend le temps de l'intervention générale et celui de l'explication de vote.

Notre discussion d'aujourd'hui est beaucoup plus politique qu'il n'y paraît : il s'agit de définir, par le truchement de la dette et de la créance, le rôle de l'État en tant qu'actionnaire et en tant

c'est-à-dire la charge de la dette, le coût que nous supportons aujourd'hui pour assumer les décisions d'hier. Il s'agit d'une ligne incontournable de notre budget : le montant de ses crédits de paiement est le troisième plus important

Or c'est précisément parce que nous avons trop longtemps cédé aux sirènes de la dette que nous ne pouvons pas saisir cette opportunité. Très bien ! Nous avons trop longtemps repoussé les réformes structurelles engagées C'est parce que nous avons manqué de sérieux budgétaire que nous avons moins de marges de manoeuvre. En laissant filer notre dette, nous avons aussi un peu renoncé à notre liberté d'action. Il y va de la résilience de notre pays face aux aléas économiques et géopolitiques. Que se passera-t-il quand les taux remonteront ? Certes, le choc sera certainement moins brutal que ce qu'annoncent les crieurs d'apocalypse, mais il est inévitable dans le temps. Il importe donc de se prémunir contre ces incertitudes qui hypothèquent notre avenir. C'est pourquoi l'augmentation de 5 milliards d'euros des crédits alloués aux dégrèvements ne constitue pas vraiment une bonne nouvelle, quand bien même il s'agit de crédits évaluatifs, et non de plafonds de dépenses. Il paraît crucial d'accélérer le désendettement de l'État. Les cessions d'actifs décidées par le Gouvernement et actées dans le cadre de la loi Pacte devraient y contribuer.

Ce choix permet d'articuler obligation de responsabilité budgétaire et nécessité d'investir dans le futur. Il est sans doute trop facile de regretter, en même temps, que le désendettement de l'État et sa stratégie d'investissements soient trop peu ambitieux. Pour le groupe Les Indépendants, il s'agit plutôt là d'alléger le poids du passé sans obérer l'avenir. Nous soutenons la mobilisation de fonds visant à financer l'innovation de rupture afin de préparer notre pays aux enjeux de demain.

trois missions qui touchent à des sujets différents et dont les budgets additionnés s'élèvent à près de 200 milliards d'euros. J'observe d'ailleurs que l'Assemblée nationale a retenu un découpage différent, ce qui témoigne de la porosité de cette discussion avec celle sur les crédits de la mission « Économie » et celle qui suivra sur le budget des administrations de Bercy et le patrimoine immobilier de l'État. Voici, en résumé, ce qui caractérisera ces différentes missions une hausse marquée des restitutions d'impôts aux particuliers et aux entreprises dans la mission « Remboursements et dégrèvements », une baisse significative de la charge de la dette dans la mission « Engagements financiers de l'État », la poursuite du Grand plan d'investissement dans la mission « Investissements d'avenir ».

que ce n'est pas à proprement parler une politique publique. Les remboursements et dégrèvements sont en hausse continue depuis plusieurs années ; l'année prochaine ne fera pas exception. Comment comprendre cette évolution ? Est-elle due à un nombre croissant d'erreurs dans le recouvrement de l'impôt ou bien à de mauvaises déclarations par les contribuables ? Notons en particulier le montant des restitutions pour le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu : 10 à 15 milliards d'euros ! Les restitutions portant sur la taxe d'habitation connaissent quant à elles la plus forte hausse-

Enfin, je suis frappé par le montant des remboursements de crédits de TVA, qui représentent la majeure partie de ce budget. Il est vrai que la TVA est la plus importante ressource de l'État. Ces remarques émises, je ne vois pas de raison de nous opposer à l'adoption de ces crédits, puisqu'ils ne sont qu'évaluatifs, mais je serais heureux de recevoir quelques éclaircissements sur les points que Je n'ai pas d'observations particulières à formuler sur les articles rattachés, qui prévoient simplement la remise de rapports. En ce qui concerne la mission « Engagements financiers de l'État la charge de la dette, portée par le programme 117, s'établit à 38,1 milliards d'euros, soit 4 milliards d'euros de moins que l'an dernier. Le passage sous la barre symbolique des 40 milliards d'euros est une bonne nouvelle de ce On ne peut toutefois pas parler de cagnotte, dans la mesure où le budget reste en déficit, et ce malgré des besoins réels dans certains domaines. Conséquence de la situation monétaire l'endettement se stabiliserait à 98,7 % du PIB, comme en 2019. C'est la première fois depuis la crise de 2008 que l'on constate une stabilisation, même si le niveau d'endettement Aussi, le besoin de financement de l'État progressera encore en 2020, mais davantage pour rembourser les intérêts de la dette passée que pour financer le déficit. Voilà donc quelques éléments d'amélioration, dans ce qui reste néanmoins le deuxième ou troisième poste de dépense. Parmi les autres budgets notables attachés à cette mission, je relève le fonds de soutien aux collectivités ayant contracté des emprunts toxiques,

autant de dispositifs dont les effets mériteraient d'être éclaircis dans un contexte de taux d'intérêt négatifs. Le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » sera marqué par les privatisations approuvées dans la loi Pacte, dont nous connaissons tous les enjeux. Après des cessions d'un montant de 8 à 10 milliards d'euros, le portefeuille de l'État actionnaire sera sensiblement réduit. L'enjeu majeur est désormais le financement et le bon fonctionnement du fonds pour l'innovation de rupture, devenu fonds pour l'innovation et l'industrie. Placé sous l'autorité de Bpifrance, il doit apporter un soutien aux projets innovants, à hauteur de 250 millions d'euros par an. Continuer à investir tout en se désendettant, voilà l'équation difficile que doit résoudre le Gouvernement. J'en viens justement à la mission « Investissements d'avenir lancement du premier PIA, voilà une décennie, par la commission Juppé-Rocard, 46 milliards d'euros ont été investis et plus de 6 000 projets ont été soutenus. Il me semble pertinent de continuer à soutenir ce budget qui finance des projets innovants, d'autant que l'investissement représente globalement une part réduite du budget de l'État. Il faut, en particulier, améliorer l'effet de levier du PIA 3, afin de le rapprocher de celui du Plan d'investissement pour l'Europe lancé par l'ancien président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui a obtenu des résultats très positifs. J'ai formulé un certain

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous devons aujourd'hui étudier les crédits de plusieurs missions et comptes spéciaux. Je ne pourrai donc être exhaustif, mais j'insisterai sur plusieurs points. La mission « Investissements d'avenir » contient des crédits qui viennent soutenir la vision d'un État stratège. Elle porte des engagements qui dépassent les clivages partisans, tant les enjeux qu'elle sous-tend sont structurants pour la croissance à venir de notre pays. Le programme d'investissements d'avenir, acté en 2010, a été relancé en 2014, puis en 2017, pour un total de 57 milliards d'euros en autorisations d'engagement.

a fait l'objet de la création de la mission que nous étudions, composée de trois programmes : « Soutien des progrès de l'enseignement supérieur et de la recherche », « Valorisation de la recherche » et « Accélération de la modernisation des entreprises

3 est désormais intégré dans le Grand plan d'investissement présenté au mois de septembre dernier, avec pour objectif de créer un choc d'offre et de doper la croissance du PIB.

empêcher des investissements privés de long terme et qui expliquent que certains secteurs ne parviennent pas à financer des projets de long terme pourtant viables du point de vue économique. Pour le dire autrement, mes chers collègues, le marché ne peut pas tout et l'intervention de l'État a, économiquement, toute sa place. Je crois d'ailleurs que le choix qui a été fait, dans le PIA 3, de structurer les priorités de l'amont vers l'aval de la chaîne de production, à partir de l'enseignement et de la recherche, et en direction de l'innovation et du développement des entreprises, se révèle utile, tant il est difficile d'identifier les nouveaux produits ou les nouvelles technologies qui émergeront à l'avenir.

Cette faiblesse des taux d'intérêt est retracée dans le programme 117 de la mission « Engagements financiers de l'État ». Selon moi, si tous les groupes politiques partagent le même souci de bonne tenue des finances publiques, nous pouvons nous réjouir que les crédits alloués à la charge de la dette et à la trésorerie de l'État aient diminué entre la loi de finances pour 2019 et le projet de loi de finances pour 2020, passant de 42 milliards d'euros à 38 milliards d'euros. d'euros. Rappelons que c'est le niveau prévisionnel le plus faible depuis 2002, alors même que l'État assume cette année la reprise de la dette de SNCF Réseau. Je crois que nous pouvons nous pouvons d'ailleurs, sans l'écarter pour autant, minorer le risque qu'une hausse des taux pourrait faire peser sur la soutenabilité de la dette publique. En effet, la France a profité de la faiblesse des taux d'intérêt pour allonger l'échéance de sa dette dette : parce que la dette publique présente aujourd'hui une maturité assez longue, une hausse des taux d'intérêt ne devrait pas se traduire immédiatement par une hausse des intérêts à verser.

Bocquet. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il est complexe d'évoquer en cinq minutes les impôts locaux, la taxe d'habitation, la retenue à la source, les crédits d'impôt, l'État actionnaire et les investissements d'avenir ! Je concentrerai donc mon propos sur l'État actionnaire.

Un tel programme de cessions, stratégiques à plusieurs titres, soulève de nombreuses questions et démontre que le Gouvernement considère que l'État est un actionnaire comme un autre fait ainsi fi d'un héritage ancien. Or, comme le soulignait la Cour des comptes en 2017, « l'État n'est pas un actionnaire comme un autre », car ses motifs de politique économique ou sociale ou de souveraineté « dépassent les seules dimensions patrimoniales « la multiplicité des objectifs poursuivis, souvent contradictoires, caractérise l'État actionnaire ». Ces contradictions sont le propre de l'État. Vouloir faire de l'État un opérateur commun, c'est dénaturer sa participation dans l'économie nous ne pensons pas que les entreprises publiques doivent être des entreprises comme les autres, car elles sont un levier majeur pour transformer l'économie et répondre aux exigences en matière d'environnement et de justice sociale. Nous ne sommes pas les seuls à le penser. Dans son rapport pour avis, Alain Chatillon rappelle que le portefeuille de l'État est avant tout un « instrument au service de la politique stratégique de l'État particulier les cessions, ne sauraient servir simplement de variable d'ajustement à la politique budgétaire conduite par le Gouvernement : la prise en compte d'enjeux industriels, de compétitivité et de souveraineté économique doit toujours primer sur la logique budgétaire. » » Nous ne pourrons peser face aux multinationales « qu'à partir d'une politique industrielle française stratégique, dont les participations financières de l'État sont une des déclinaisons

Il en va de même de la privatisation d'Aéroport de Paris (ADP), qui reste un actif stratégique, quoi qu'en pense le Gouvernement. Je rappelle que la valorisation boursière de ce groupe a été multipliée par quatre en dix ans, dans un contexte où le transport aérien devrait encore fortement croître au cours des prochaines années.

Le pire est que le Parlement est dessaisi : il n'intervient pas sur l'évolution de ce portefeuille. Certes, il doit se prononcer sur les privatisations en tant que telles, mais il ne peut pas participer à la définition de la stratégie actionnariale de l'État. De même, il ne peut se prononcer sur les mouvements financiers, en d'autres termes les achats et les ventes de titres. Comme le soulignait la rapporteure à l'Assemblée nationale, le Parlement n'a aucun pouvoir non plus sur l'affectation des dividendes issus des participations de l'État,

La mission « Remboursements et dégrèvements » constitue, en volume, la plus importante du budget général de l'État : les crédits ouverts s'établiront à 141 milliards d'euros en 2020, soit le tiers des recettes fiscales brutes et près de la moitié des recettes nettes. Ils représentent une hausse de 6 milliards d'euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2019. Dans les grandes masses, cette augmentation s'explique, malgré le recul des dépenses contentieuses,

J'en viens aux crédits de la mission « Engagements financiers de l'État », destinés à assurer le financement de l'État en toutes circonstances, à garantir ses positions liées au développement international de l'économie française et à favoriser les politiques d'épargne. mission couvre presque exclusivement la charge de la dette publique, qui représente 99 % de ses crédits. La dette française atteindrait ainsi 98,7 % du PIB à la fin 2020, soit plus de 40 points de plus que l'Allemagne l'an prochain et près de 40 points de plus que notre propre ratio

Nous pourrions nous féliciter de la baisse des crédits de la mission, qui sont en reflux de 4 milliards d'euros, d'autant plus qu'elle résulte principalement de la diminution de la charge de la dette. celle-ci n'est que la conséquence de taux d'intérêt extrêmement favorables, nullement le fruit d'efforts consentis par notre pays en faveur de la réduction de la dépense et du désendettement publics. D'ailleurs, la dette de l'État, en valeur nominale, est en nette augmentation, puisqu'elle devrait passer de 1 806 milliards d'euros en 2019 à 1 891 milliards d'euros en 2020. C'est une charge terrible qui est ainsi transmise aux générations futures, sur les épaules desquelles

financé par la dette. Cela signifie concrètement que l'impôt aujourd'hui sert non pas à résorber l'endettement de l'État, mais à financer de nouvelles dépenses, en plus de celles qui sont déjà prévues. Non seulement nous vivons à crédit, sur les dépenses des générations futures, mais, au surplus, nous obérons notre capacité d'investissement public. Dans un contexte marqué par l'incertitude géoéconomique et géostratégique et par des perspectives de croissance pour le moins dégradées, il est urgent d'engager un réel effort structurel de désendettement, afin que soit tenu l'objectif fixé par le Gouvernement d'une réduction de la dette publique à hauteur de 5 points de PIB. Il s'agit tout à la fois de nous préserver de toute difficulté en cas de remontée soudaine des taux d'intérêt, de nous ménager d'indispensables marges de manoeuvre et, de façon moins moins anecdotique qu'on ne le croit, de respecter les engagements pris devant les Français par le Président de la République au début du quinquennat. Je dirai enfin un mot sur la mission « Investissements d'avenir ». Le programme d'investissements d'avenir, qui est aujourd'hui en phase 3, constitue un soutien public de 10 milliards d'euros à l'enseignement supérieur, à la recherche et à la modernisation des entreprises. Si nous ne pouvons que nous réjouir de l'objectif affiché, nous demeurons vigilants, je tiens à le redire ici, sur les évaluations qui doivent être conduites en la matière.

La dette, qu'avec respect tout le marché admire, « La dette, qui a tant de fois sauvé cet empire, « Trahit donc ma querelle, et ne fait rien pour moi ? » Voilà ce qui risque d'arriver si nous

Cette hausse globale de 1,68 % recouvre des variations, dont les causes sont diverses. Vos explications seraient les bienvenues à cet égard, monsieur le ministre.

Les remboursements et dégrèvements liés à la taxe d'habitation, qui s'élèvent désormais à 14,7 milliards d'euros, constituent la majeure partie de la dépense, manifestement du fait de la réforme de la taxe d'habitation. Ainsi, Ainsi, ces remboursements et dégrèvements devraient représenter un tiers environ des recettes fiscales brutes correspondantes. Cette proportion, en constante augmentation, met en évidence que la politique fiscale repose essentiellement sur des décisions de nature à grever les ressources de l'État et à entraver ses marges d'action. Un réexamen des choix politiques qui sous-tendent ces évolutions nous semble d'évidence justifié. Au regard de ces éléments globaux et malgré les réticences que je viens d'exprimer concernant notamment les orientations politiques du Gouvernement,

avec un total de 38 145 milliards d'euros pour 2020, soit une baisse de 9,3 %. Cette situation s'explique mécaniquement par la baisse des taux d'intérêt et par les taux négatifs, qui allègent la charge de la dette pour Bien qu'il y ait évidemment lieu de se réjouir de cet état de fait positif pour les finances publiques, nous ne devons pas nous laisser gagner par une euphorie anesthésiante ! Vous le savez, mes chers collègues, la faiblesse actuelle des taux est atypique et nul ne peut raisonnablement prédire combien de temps elle durera.

La mission « Investissements d'avenir » retrace les crédits du troisième programme d'investissement (PIA 3), adopté en 2017 et doté de 10 milliards d'euros pour la période 2018-2022. Pour 2020, les crédits demandés s'élèvent à 2,18 milliards d'euros, alors que le montant initialement inscrit était de 1,88 milliard d'euros. Le Gouvernement s'écarte donc de la trajectoire budgétaire du PIA 3, puisqu'il dépasse le plafond de 4 milliards d'euros prévu sur la période triennale 2018-2020.

En dépit d'une hausse apparente de plus de 43 % du programme, les crédits de paiement à destination des opérateurs de l'État sont néanmoins en baisse. En effet, l'Agence nationale de la recherche a reçu 185 millions d'euros en 2019, alors que 115 millions d'euros sont prévus pour 2020. (Ademe) est également affectée, le projet de loi de finances pour 2020 prévoyant de lui accorder 37 millions d'euros en crédits de paiement, contre 40 millions d'euros antérieurement. antérieurement. Les deux opérateurs chargés d'atteindre les deux objectifs du programme- faciliter l'approche de l'innovation et soutenir les investissements concourant au renforcement de la performance environnementale dans le parc industriel -voient leurs moyens diminuer par rapport à l'exercice antérieur.

Enfin, le CAS « Participations financières de l'État » contribue au désendettement à hauteur de 2 milliards d'euros, soit une goutte d'eau au regard des besoins. D'ailleurs, notre rapporteur spécial estime que cet argent pourrait être mieux utilisé pour soutenir les entreprises du portefeuille de l'État.

Le programme 117, « Charge de la dette et trésorerie de l'État », et le programme 731, « Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État », contribuent tous deux à alimenter le fonds pour l'innovation et l'industrie. Le contrôle du Parlement sur ce fonds est faible, ce dernier étant géré par le Conseil de l'innovation. La Cour des comptes a d'ailleurs formulé des critiques justifiées dans une note d'exécution budgétaire récente : ce fonds permet « une affectation directe, en dehors du budget de l'État, de recettes de cessions de titres et de dividendes pour réaliser des actions qui auraient pu être financées par des programmes budgétaires ». Les 25 millions d'euros versés par fonds de concours au programme 120 dans le projet de loi de finances Les crédits du PIA sont difficiles à suivre, car ils sont ventilés sur un grand nombre d'actions, ces dernières étant mises en oeuvre par quatre opérateurs. Le Parlement dispose également de peu de moyens pour contrôler les engagements hors bilan, dont le volume a été multiplié par trois ces dernières années. années. Depuis 2013, les restitutions de TVA ont augmenté de plus de 11 milliards d'euros. Le mouvement se poursuit en 2020, les restitutions prévisionnelles étant supérieures de 3,5 % au montant de 2019 actualisé. Le Parlement demande à être mieux informé sur le niveau de la fraude à la TVA, compte tenu de l'enjeu pour les finances publiques. Dans son référé du mois de décembre 2018, la Cour des comptes relevait que les indicateurs spécifiques à la délinquance économique et financière, qui figuraient dans les projets et les rapports annuels de performance des programmes 152, « Gendarmerie nationale », et 176, « Police nationale », de la mission « Sécurités », avaient disparu depuis 2014. 2014. Ces missions et ce CAS présentent des zones de risques. Les conditions de rémunération de la dotation en numéraire du fonds pour l'innovation et l'industrie sont strictement supérieures à ce qui s'observe sur les marchés, ce qui laisse augurer des lendemains douloureux lors de la clause de revoyure fixée à 2023. Par ailleurs, année après année, les prévisions du programme 200, « Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État », demeurent inférieures aux coûts potentiels des contentieux de droit de l'Union européenne, lesquels se chiffrent à plus de 10 milliards d'euros. à plus de 10 milliards d'euros. Enfin, l'encours de dette négociable est en hausse constante ces dix dernières années. Cet accroissement traduit l'incapacité de l'État à assainir ses finances publiques. En cas de remontée des taux, la charge de la dette pourrait être multipliée par 1,5 en moins de dix ans.

comme pour les taux bas. La prévision pour 2020 fait l'hypothèse- prudente -que le taux à 10 ans est amené à rebondir légèrement, depuis les plus bas historiques atteints à l'été 2019. Le taux à 10 ans s'élèverait à 0,20

la charge de la dette atteindrait 38,6 milliards d'euros en 2020, soit un niveau inférieur de 1,9 milliard d'euros à la prévision actualisée pour 2019, comme l'a notamment souligné Guillaume Arnell.

d'euros les deux années suivantes. Pour continuer de bénéficier de taux d'intérêt favorables, il est important de garder la confiance des investisseurs en ne déviant pas de la trajectoire de consolidation des finances publiques. Cette situation doit nous inviter à poursuivre les réformes structurelles pour maîtriser les déficits publics. À cet égard, le Gouvernement est résolu à maîtriser la dépense publique,

La profonde modernisation engagée au sein de la direction générale des entreprises permettra en particulier d'économiser 152 emplois. Hors charge de la dette, les autres engagements financiers de l'État sont maîtrisés, grâce à des actions engagées par le ministère. Je citerai ici l'assurance prospection. Géré depuis 2017 par Bpifrance Assurance Export, et réformé en 2018, ce dispositif offre aujourd'hui à 11 000 PME une assurance contre le risque d'échec des actions de prospection à l'étranger, en prenant en charge une part des frais non amortis par un chiffre d'affaires suffisant sur la zone concernée.

nous nous donnerions les moyens de respecter l'engagement de la France pour la rétrocession des intérêts perçus sur le capital placé auprès des institutions européennes. La programmation retenue pour le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » témoigne, elle aussi, de notre volonté de maîtriser les finances publiques tout en disposant de marges de manoeuvre pour soutenir l'innovation.

qui justifie l'inscription de crédits notionnels. Les réflexions actuelles portant sur les modalités de mise en oeuvre de la LOLF conduiront vraisemblablement à revisiter la construction et le suivi des indicateurs de performance associés aux différentes politiques publiques. Dans ce cadre, le ministère saisira toute occasion de répondre

par ses conditions de mise en oeuvre, il offre des modalités de soutien uniques. La réintégration du FII dans le budget général n'est pas pertinente à ce stade : il convient de garantir la stabilité des dispositifs, gage de confiance pour les acteurs économiques, et leur souplesse d'utilisation, qui est essentielle à une mise en oeuvre efficace des actions proposées. Je terminerai en abordant les questions qui ne relèvent pas directement du ministère de l'économie et des finances. Monsieur Savoldelli, l'évolution des demandes de remboursement de TVA déposées par les entreprises auprès des services de la direction générale des finances publiques est liée à celle de certains agrégats macroéconomiques. Ainsi, lorsque leurs investissements ou leurs consommations intermédiaires les entreprises sont davantage en situation de crédit. Par ailleurs, le coût des contentieux fiscaux est, pour une part, le reflet de la sollicitation accrue des tribunaux par les contribuables et du développement de contentieux de masse. Il résulte également de la complexité de la norme fiscale. Ces constats

Il s'agit de consacrer un effort d'investissement exceptionnel, ciblé sur les projets les plus structurants et prometteurs, au-delà des actions poursuivies par les ministères dans le cadre budgétaire habituel. Le fonctionnement de ce programme repose sur des procédures de sélection ouvertes et compétitives, au moyen d'une stratégie interministérielle et transparente.